La séance est reprise.

de la société civile, tous canaux confondus, pour atteindre 620 millions d'euros en 2022. Compte tenu de la situation économique pour le moins incertaine, il ne paraît pas opportun d'inscrire dans ce projet de loi une cible nominale. La marche à franchir pour atteindre 1 milliard d'euros nous semble, en l'état de la trajectoire des crédits du programme 209, inatteignable en trois Messieurs les rapporteurs, vous avez évoqué les risques inhérents à une APD trop rigide et impossible à piloter. Nous sommes précisément en présence d'un tel risque : cumuler des contraintes sur la concentration géographique et sectorielle, d'une part, et sur les canaux, canaux, d'autre part, reviendrait à rigidifier à l'extrême le pilotage global de l'APD. La parole

Il s'agit ainsi de mentionner explicitement que l'État associe à la politique de développement solidaire les organisations de la société civile française et des pays partenaires, les destinataires des actions de développement solidaire, les citoyens engagés, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, ainsi que les partenaires sociaux. préciser que le Gouvernement instaure un dialogue annuel avec eux.

Guillaume Gontard. Cet amendement vise à compléter le dispositif de base de données ouvertes regroupant les informations relatives à l'aide publique bilatérale et multilatérale de la France, qui a été ajouté à l'Assemblée nationale et dont nous nous réjouissons.

soutiens qui contribuent à son influence à l'étranger. Cela permettrait d'avoir une vision complète de la politique d'aide publique de la France et de sa cohérence. Ensuite, à des fins de lisibilité et d'exhaustivité, cette base de données doit inclure les budgets totaux, les budgets désagrégés, les rapports de résultats et les évaluations des soutiens financiers hors APD octroyés par l'État, ses opérateurs et l'ensemble des établissements publics et semi-publics participant à l'action extérieure de la France dans les pays en développement, notamment Proparco et Bpifrance. Pour les mêmes raisons, nous proposons également d'y inclure les analyses des impacts sociaux et environnementaux de l'APD française et des autres soutiens français. À ce jour, ces flux financiers ne font pas l'objet de transparence, alors que l'action de l'APD souffre déjà d'un sérieux manque de lisibilité et que ces flux ont une incidence majeure sur le modèle de développement que suivent ces pays. La transparence et la redevabilité de l'APD sont pourtant indispensables à l'approche partenariale qui est promue par le texte que nous examinons aujourd'hui. En commission, les rapporteurs nous ont opposé le fait que cette base de données était trop exhaustive, donc potentiellement excluante.

leurs filiales et les établissements publics et parapublics marquerait une volonté de transparence. Le groupe CRCE s'est toujours battu et continuera à se battre pour mettre fin au transit de fonds publics de l'aide au développement vers des paradis fiscaux. Rappelons-nous que, le 11 juin 2014, a dévoilé comment la filiale de l'AFD, Proparco, avait investi plus de 400 millions d'euros dans des sociétés situées à l'île Maurice, aux îles Caïmans et au Luxembourg, véritable enclave fiscale au sein de l'Europe. Nous réaffirmons ici que cet investisseur privé agit pour le compte de l'État et ne peut être mû par des objectifs de rentabilité au détriment de l'intérêt général et des bonnes pratiques en matière fiscale. Certes, l'AFD s'est dotée en 2016 d'une liste de juridictions non coopératives dans laquelle figurent 14 États, mais le problème d'une liste, c'est souvent ce qu'elle ne contient pas ! Ainsi ne sont pas considérées comme des paradis fiscaux la République de Malte, les îles Caïmans ou encore l'île Maurice.

Richel Group, identifiée pour fournir les serres dans le projet de Spayka. Au total, ce sont 23,5 millions d'euros que la France a engagés pour un projet allant à l'encontre de ses priorités stratégiques en matière de modèle agricole, ce dont nous n'aurions pas eu connaissance sans une enquête des ONG. Élargir le périmètre de la base de données permettrait de pallier ce manque de transparence, donc de redevabilité, pour les soutiens financiers hors APD, et de mieux affirmer l'approche partenariale de la politique de développement que nous promouvons par ce texte. Voter cet amendement est le minimum indispensable pour conférer à cette base de données une portée suffisante.

compréhensible par tous et utilisable pour le contrôle de la politique d'aide publique au développement. Si ces recommandations étaient adoptées, elles seraient aussi utiles au travail de contrôle des parlementaires

notamment ceux qui ne peuvent pas faire l'objet d'une restitution, devrait participer directement au renforcement des systèmes fiscaux des pays en voie de développement. C'est une question sur laquelle nous revenons

qui a pour inconvénient de prendre un temps non négligeable et d'empêcher l'intégration d'un bien immobilier doté d'une véritable utilité dans le patrimoine de l'État en question. Il s'agit donc d'un amendement de bon sens et de simplification, qui vise à donner un peu de souplesse à ce processus de restitution des biens mal acquis, et ce au bénéfice des populations.

un nouvel alinéa à l'article 1afin notamment de définir le champ infractionnel des biens mal acquis concernés par le nouveau mécanisme de restitution.

qui sera placé sous la responsabilité du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, et dont les modalités permettront au Parlement, et plus largement à la société civile, d'assurer chaque année le suivi de la mise en oeuvre de la restitution des biens mal acquis en autorisant, puis en contrôlant l'emploi des crédits ouverts à cette fin. Elles permettront aussi de s'assurer au mieux de la transparence et de la redevabilité du dispositif. Le Gouvernement a, par ailleurs, sous-amendé l'amendement du rapporteur à l'Assemblée nationale pour mettre en place le dispositif proposé. Les produits de cessions donneront ainsi lieu à des ouvertures de crédits au sein de la mission « Aide publique au développement ». Tout cela me paraît cohérent

Dans le même temps, cette crise fait ressortir les inégalités structurelles qui existent dans tous les domaines, depuis la santé et l'économie jusqu'à la sécurité et la protection sociale. En période de crise, lorsque les ressources s'amenuisent et que les capacités institutionnelles sont mises à rude épreuve, les situations auxquelles les femmes et les filles sont confrontées ont des impacts disproportionnés, et leurs effets sont encore amplifiés dans les contextes fragiles de conflit ou d'urgence. Les acquis arrachés de haute lutte en matière de droits des femmes sont ainsi menacés. Pour illustrer mon propos, je rappelle que les femmes sont les plus touchées par la crise économique, parce qu'elles gagnent moins que les hommes, qu'elles constituent la majorité des familles monoparentales et qu'elles sont surreprésentées dans le secteur informel. cette pandémie n'entraîne un recul de 25 ans en matière de droits des femmes. Cet amendement vise donc à faire reconnaître l'impact particulier de la crise du covid-19 sur les femmes.

la pandémie amplifie les inégalités existantes, notamment celles qui concernent les femmes. Le texte actuel mentionne déjà de façon générale l'accroissement des inégalités, mais nous n'avons pas d'objection à cet ajout. La commission émet donc un avis favorable

1 A sur l'énumération du triptyque d'objectifs principaux de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, et sur le fait que l'insécurité alimentaire constitue une dimension de la pauvreté. Il tend aussi à se conformer à la définition onusienne des biens publics mondiaux, En effet, d'après la définition du programme des Nations unies pour le développement de 1999, trois grandes catégories composent les BPM : ceux qui sont naturels,

Par conséquent, il serait préférable de citer l'éducation et la santé parmi les biens publics mondiaux. Enfin, il s'agit de faire figurer la lutte contre la pollution, qui constitue un défi majeur pour la protection de la planète, parmi les objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.

est à Mme Nicole Duranton. Cet amendement de repli vise à se conformer à la définition onusienne des biens publics mondiaux. En effet, d'après la définition du programme des Nations unies pour le développement de 1999, trois grandes catégories composent les BPM : ceux qui sont naturels tels que le climat ou la biodiversité, ceux qui sont d'origine humaine, enfin, ceux qui résultent de politiques globales, comme la paix, l'éducation et la santé. Par conséquent, il serait préférable de citer l'éducation et la santé parmi les biens publics mondiaux. Duranton. Cet amendement de repli a pour objet de faire figurer la lutte contre la pollution, qui constitue un défi majeur pour la protection de la planète, parmi les objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. L'amendement Lepage. L'égalité entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs paragraphes du cadre de partenariat global et est désormais introduite dans le corps du texte, ce qui constitue une avancée par rapport au projet de loi initial. Toutefois, sortie de ces paragraphes particuliers, l'égalité entre les femmes et les hommes n'a plus d'existence, alors que sa transversalité et la nécessité qu'elle irrigue tous les champs d'action de l'aide publique au développement doivent être au coeur de notre politique. La France revendique une diplomatie féministe. Cette politique à visée transformative implique un changement de paradigme dans l'ensemble des dimensions de notre politique extérieure.

Pour cela, il préconisait que le périmètre défini englobe tous les domaines de la politique étrangère. Les droits des femmes sont encore trop souvent considérés comme une simple thématique.

Pourtant, n'est-ce pas cette vision qui prévaut lorsque Florence Parly, auditionnée au début de l'année 2019 par la commission des affaires étrangères du Sénat, affirme que « pour se prémunir autant que possible contre le risque de rejet de la présence militaire étrangère, il faut aussi mener des projets de développement armées d'ajouter : « À cet égard, nous souhaitons articuler de manière plus efficace l'action de Barkhane et les actions de l'Agence française de développement, pour que le rétablissement de la sécurité bénéficie directement aux populations. C'est ainsi que la présence militaire sera mieux tolérée Ces propos accréditent, aux yeux d'un nombre croissant d'acteurs, que l'AFD est finalement utilisée comme un masque derrière lequel se cache l'armée française. Le développement ne doit pas rester le troisième « D » enfermé dans la stratégie dite des 3D : défense, diplomatie, développement. Il ne peut pas être l'alibi d'une stratégie militaire et diplomatique dans l'impasse, il doit être l'ambition autour de laquelle tout doit s'organiser. Permettez-moi également d'évoquer le fait que la France tient, de fait, le stylo en ce qui concerne les résolutions de l'ONU traitant des pays de son pré carré. nous ne sommes pas hostiles aux appuis militaires dans le cadre des Nations unies, nous gardons à l'esprit cet état de fait, qui jette souvent un doute sur ceux-ci., nous ne pouvons considérer que la coopération militaire participe au champ de l'APD. Pour mettre un terme à cette confusion, mes chers collègues, je vous invite à adopter cet amendement, qui vise à sortir la coopération militaire de la France du champ de l'APD. Quel

16 nous appelle à apporter collectivement une réponse coordonnée aux défis rencontrés par les pays bénéficiaires en améliorant l'articulation et la cohérence des actions des différents acteurs relevant de la défense, de la sécurité, de l'humanitaire et du développement. Il existe parfois des logiques divergentes, mais il faut assurer la cohérence de

établie le 10 décembre dernier par le bureau du conseiller spécial pour l'Afrique de l'ONU, laquelle pose d'autres enjeux de sécurité dont nous ne nous occupons pas assez. C'est le cas, par exemple, des flux financiers illégaux

de ce document, l'un des objectifs centraux, s'appuyant d'ailleurs sur la feuille de route de Lusaka de 2016, est la suppression des paradis fiscaux offshore qui sont utilisés

définit les grands objectifs et principes d'action de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. L'alinéa 12 indique que celle-ci concourt à la politique étrangère de la France ainsi qu'à son rayonnement et à son influence culturelle, diplomatique et économique. L'influence sportive de la France n'est malheureusement pas prise en compte. L'objet de cet amendement est donc de remédier à cet oubli. Le sport est spécifiquement mentionné dans la déclaration des Nations unies sur les objectifs de développement durable. Les mouvements olympiques et paralympiques internationaux s'inscrivent également dans cette démarche.

pour présenter l'amendement n° 230. Le cadre de partenariat global fixe les objectifs principaux de notre politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Parmi ceux-ci figure la promotion des droits de l'enfant. Pour autant, le respect et la promotion des principes et des normes internationaux en matière de droits de l'enfant ne sont pas prévus. Comme l'a souligné ma collègue, dans le cadre de la loi de 2014, les principes directeurs de la Convention internationale des droits de l'enfant étaient pourtant mentionnés expressément. Ce projet de loi ne les reprend pas, alors même que la ratification de la Convention internationale des droits de l'enfant, intervenue en 1990, implique le respect et la promotion de ses principes directeurs. Cet amendement vise donc à mettre en application les engagements de la France en matière des droits de l'enfant et à prévoir leur respect et leur promotion. Quel est l'avis de la commission ? La

Cet amendement vise à remplacer la référence aux droits de l'homme par une référence aux droits humains. L'utilisation des termes « droits de l'homme » n'est pas un détail sémantique sans importance. Cette appellation n'est pas neutre, elle s'inscrit dans une histoire française qui a longtemps exclu et « invisibilisé » les femmes. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans laquelle s'enracine l'utilisation persistante de droits de l'homme en France, loin d'être universelle, excluait explicitement les femmes et a longtemps permis de les écarter du droit de vote et de la vie politique. Jamais, il n'a été dans l'intention des auteurs de la déclaration de 1789 d'accorder aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes. Je n'ai pas besoin de rappeler ici l'action d'Olympe de Gouges Par ailleurs, l'expression « droits de l'homme » isole la France. La plupart des pays européens utilisent « droits humains ». Il n'est évidemment pas question de modifier le titre de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui font partie intégrante de notre histoire, s'agit de privilégier l'expression « droits humains » pour tout autre usage, afin d'en finir avec la logique discriminatoire encore véhiculée par la langue française.

Compte tenu des multiples références aux droits des enfants introduites dans le texte et l'importance de cette population dans de nombreux pays en développement, la commission émet un avis favorable

instruments et engagements pris par la France en matière de droits des femmes doivent être diffusés par le biais de notre politique d'aide publique au développement. C'est d'autant plus vrai en matière de droits des femmes, puisque les cadres multilatéraux afférents font l'objet de nombreuses attaques ou critiques. Le retrait de la Turquie de la convention d'Istanbul par un simple décret présidentiel au mois de mars 2021 en est un exemple criant. Pour rappel, seuls trente-trois pays sur les quarante-sept États membres du Conseil de l'Europe l'ont ratifiée, et la Pologne semble se diriger à son tour vers une dénonciation. Cet épisode pourrait être le signe avant-coureur d'un mouvement plus large de dénonciation des instruments de protection des droits fondamentaux. Afin d'éviter cela dans notre pays affirmer les valeurs françaises, cet amendement vise à inclure la convention d'Istanbul, la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, également attaquée par les milieux conservateurs turcs, et la déclaration et le programme d'action de Beijing dans le cadre général de mise en oeuvre de notre politique d'aide publique au développement.

proposée tend à insérer la convention d'Istanbul, parmi d'autres, dans un paragraphe dédié au cadre multilatéral onusien. Or il s'agit d'une

dans le cadre de la lutte contre les inégalités mondiales, les recommandations de l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Il est bien

le CPG toute une série de conventions et d'accords internationaux dont la France est partie prenante risque de faire catalogue.

Alors que l'on observe certaines avancées importantes, quoiqu'inégales, dans la promotion des droits des femmes et des filles, aucun pays au monde ne semble actuellement en bonne voie pour parvenir à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et à l'émancipation de toutes les femmes et filles à l'horizon 2030. De plus, les effets sanitaires et socioéconomiques de la crise de la covid-19 touchent actuellement les femmes et les filles de manière disproportionnée. Ainsi, étant donné qu'une plus grande proportion de femmes occupe un emploi informel en travaillant dans des secteurs vulnérables, le rythme des suppressions d'emplois les concernant est 1,8 fois supérieur à celui des hommes. Le taux de pauvreté parmi les femmes pourrait s'élever à 9,1 %. Pour y remédier, le nouveau plan d'action de l'Union européenne sur l'égalité des genres et l'émancipation des femmes dans l'action extérieure 2021-2025 vise à accélérer les progrès en matière d'émancipation des femmes et des filles, tout en sauvegardant les gains réalisés en matière d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long des vingt-cinq années ayant suivi l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Pékin. Ce troisième plan d'action dote l'Union européenne d'un cadre stratégique s'articulant autour de cinq axes d'action qui visent à accélérer les progrès nécessaires au respect des engagements internationaux et à faire en sorte que le monde offre à chacun la possibilité de s'épanouir. Ce plan fait de la promotion de l'égalité une priorité de toutes les politiques et actions extérieures et prévoit une feuille de route pour travailler conjointement avec les parties prenantes à l'échelon national, régional et multilatéral. Il intensifie l'action dans des domaines thématiques stratégiques. Il appelle les institutions à montrer l'exemple et garantit la transparence des résultats. Véritable pilier de l'action extérieure de la France, le plan d'action Genre de l'Union européenne doit être cité comme partie prenante du cadre de partenariat global de mise en oeuvre de notre aide publique au développement.

2021 à 2025 et n'est pas du même niveau normatif qu'une convention internationale. Il est par ailleurs fait référence à ce plan dans le chapitre du CPG consacré à la priorité transversale de l'égalité entre les femmes À mon avis, il n'est pas pertinent d'inclure une référence à ce plan d'action dans cet alinéa qui vise à rappeler que la politique de développement de la France s'inscrit dans le cadre européen, notamment dans le consensus européen pour le développement de 2017. Il y a un défaut de méthode

continents et sur les trois grands océans. Les collectivités, départements et territoires d'outre-mer sont une richesse pour notre pays et un atout

l'importance de l'action extérieure des collectivités d'outre-mer dans leur bassin régional, en particulier en matière de coopération et de développement. Vous le savez, nos opérateurs peuvent

Cet amendement a pour objet de permettre aux TPE-PME de droit local détenues par des entrepreneurs français à l'étranger (EFE) ainsi qu'aux filiales de TPE-PME françaises à l'étranger de bénéficier d'un accès facilité au crédit par le biais de garanties offertes par l'AFD. Je pense, comme nombre de nos collègues, que la France doit reconnaître le rôle actif des entrepreneurs français à l'étranger comme vecteur de l'efficacité de notre politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Je me suis rendu en Équateur, à Manta, trois ans après le tremblement de terre de 2016, qui avait fait plus de 1 000 victimes. J'y ai rencontré des entrepreneurs français qui avaient tout perdu : qui une usine de purification d'eau, qui un élevage de crevettes avec des bassins sur 100 hectares, j'en passe. Ces compatriotes déploraient que la France ne leur ait offert aucune assistance pour faciliter le redémarrage de leurs activités. Si tous saluaient l'intervention de la France, notamment pour approvisionner en eau potable les villes touchées par le séisme, ils voulaient savoir pourquoi ils ne pouvaient, quant à eux, prétendre aux aides apportées par l'AFD. Le covid s'est révélé être un séisme mondial pour les entrepreneurs français à l'étranger. Dès le début de la crise, j'avais évoqué le dispositif Harris destiné à créer un mécanisme d'urgence pour appuyer le redémarrage de petites structures.

L'aide publique au développement doit également être plus agile et permettre à nos TPE-PME de se relever au plus vite lorsqu'elles sont confrontées à des circonstances exceptionnelles. Quel est l'avis de

important dans le tissu économique local des pays partenaires. Il est donc pertinent de rappeler que l'AFD ou Proparco, par le biais des garanties offertes dans ces pays, peuvent faciliter leur accès au crédit en cas de circonstances exceptionnelles. La commission émet un avis favorable sur cet amendement. Quel est

souhaitez que l'aide au développement intègre l'encouragement à la réalisation de projets par des entreprises françaises installées à l'étranger. Or c'est contraire aux normes de l'OCDE, je me permets de vous le rappeler,

Conway-Mouret. Le Président de la République a, dès le début de son quinquennat, exprimé sa volonté de placer la diaspora au coeur de la dynamique nouvelle qu'il entend donner aux relations franco-africaines, en vue d'impulser un réel développement allant dans le sens de nos intérêts communs. Si cette initiative est bienvenue, elle ne doit en aucun cas relever d'un simple effet d'annonce. Il est nécessaire d'aller plus loin en renforçant les actions des diasporas, afin de faire d'elles des actrices du développement bénéficiant d'une reconnaissance officielle. En effet, les diasporas représentent une véritable richesse. D'une part, grâce à leur double appartenance, elles sont au croisement de plusieurs cultures et sont non seulement des ambassadrices de la France en Afrique, mais, inversement, de l'Afrique en France.

Leurs actions ont permis de doter des pans entiers de villages et de localités d'infrastructures nécessaires au développement local, telles que des écoles, des centres de santé ou encore des réseaux d'eau potable et d'assainissement. Elles sont souvent les acteurs locaux de la mise en oeuvre d'actions de coopération décentralisée, que certains d'entre nous connaissent très bien ici. Enfin, elles sont à l'origine d'importants transferts de fonds, qui sont devenus une source non négligeable de financements extérieurs pour les pays en développement. Au vu du rôle qu'elles assument déjà, l'AFD pourrait renforcer son concours apporté aux associations dans le cadre du dispositif du Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations (Forim), en vue de créer une réelle coopération fructueuse. Or, aujourd'hui, les fonds alloués à l'AFD en faveur du Forim ne sont pas prioritairement orientés vers les pays de l'Afrique subsaharienne. Il s'agirait donc d'augmenter le nombre de projets subventionnés par l'AFD en faveur du Forim, en veillant à accorder une priorité particulière aux zones géographiques définies comme prioritaires dans le cadre de l'APD de la France. Mes chers collègues, voter cet amendement est un moyen de placer les diasporas au coeur des relations franco-africaines, lesquelles gagneraient à être renforcées.

La pandémie que nous traversons a démontré à la fois la nécessité pour les États d'être autonomes dans le domaine de la recherche et l'importance d'être unis et solidaires dans le cadre de la mondialisation et de nos interdépendances. Or les pays en voie de développement, notamment ceux d'Afrique subsaharienne, manquent de matériels, tels que les outils informatiques, et de ressources humaines. Pour pallier ces difficultés, cet amendement vise à faire de l'APD de la France un instrument au service de l'essor de l'enseignement supérieur et de la recherche au sein des pays bénéficiaires, afin de favoriser leur autonomie dans ces domaines. Cela passe par des moyens pour l'achat de matériel indispensable pour la recherche et par l'accompagnement à la formation des chercheurs dans le cadre de partenariats mutuellement bénéfiques. Cette disposition s'inscrit dans la volonté de développer des laboratoires de recherche dans les pays en voie de développement et de donner aux chercheurs les moyens d'y conduire leurs travaux.

et dans l'ouverture de la jeunesse à l'international, au travers d'échanges et de projets internationaux. La mention explicite du rôle du sport sera un point d'appui utile pour développer et renforcer les initiatives internationales, ainsi que pour atteindre ces objectifs.

D'une part, en effectuant un volontariat au sein d'entreprises ou d'organisations françaises, qu'elles soient implantées sur leur territoire ou en France, ces bénévoles peuvent acquérir des savoir-faire et des compétences et, réciproquement, relayer l'expertise française de retour dans leur pays si leur expérience a eu lieu en France. D'autre part, cette réciprocité permet de renforcer la coopération entre la France et les pays en développement, les liens entre les jeunesses du Nord et du Sud ainsi que les connexions entre les entreprises françaises et les entreprises de ces pays. Il s'agit d'un véritable facteur de fluidification des échanges dans le cadre des relations bilatérales. La France, parce qu'elle est l'un des principaux bailleurs de la francophonie, pourrait d'ailleurs s'appuyer sur une coopération avec des institutions telles que l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), notamment en renforçant le dispositif préexistant du volontariat international de l'OIF, afin de favoriser l'arrivée de volontaires originaires de pays en voie de développement. Mes chers collègues, adopter cet amendement, c'est faire le choix du développement humain, du rayonnement de la France et de son savoir-faire au travers de l'apprentissage des jeunes, tout en s'appuyant sur un bien commun, celui de la culture francophone. Cela permet surtout s'apporter des précisions sur les notions de volontariats réciproques et de mobilité croisée figurant à l'alinéa 134 projet de loi : « Dans le cadre de la trajectoire ascendante de l'aide publique au développement, l'État encourage le développement quantitatif et quantitatif et qualitatif du volontariat dans le cadre d'autres dispositifs de volontariat international existants. Il consolide le cadre de la mobilité croisée et les volontariats réciproques ... » Il s'agit donc d'entrer dans le détail d'une présentation somme toute assez vague. Quel L'article 6 élargit le volontariat de solidarité internationale pour permettre le volontariat réciproque. Le service civique est également ouvert, marginalement il est vrai, à un dispositif de volontariat réciproque. S'agissant des autres types de volontariat, l'article 12 prévoit un rapport présentant la stratégie de la France en matière de mobilité internationale au sein d'entreprises et d'administrations, concernant notamment l'opportunité d'un élargissement des conditions d'accès aux volontariats internationaux prévues par le code

fait de distinction entre le volontariat associatif, le bénévolat, les volontaires internationaux en entreprise et les volontaires internationaux en administration.

il nous paraît important de préciser ce que nous attendons des pays partenaires : le respect de l'État de droit, des droits humains et la protection des populations. Nous souhaiterions voir ces précisions figurer dans ce Quel est l'avis de la commission ? Il ne serait pas pertinent d'énumérer de manière limitative la notion de réciprocité. La réciprocité ne donne pas nécessairement lieu à des demandes précises. La politique de développement solidaire peut renforcer l'influence de la France, y compris dans les pays destinataires, et il convient de garder ouvertes les différentes modalités selon lesquelles cette influence est amenée à se traduire. La commission émet donc un avis défavorable

exhaustif le paragraphe du rapport annexé relatif à l'objectif de cohérence recherché entre la politique de développement et les politiques publiques françaises susceptibles d'avoir un impact sur les objectifs de développement durable, les ODD, en y ajoutant les politiques agricoles et alimentaires. Aujourd'hui, le discours tenu dans le CPG au sujet de l'agriculture durable est enthousiasmant. Nous affirmons ainsi que « la France promeut une agriculture familiale, productrice de richesses et d'emplois, respectueuse des écosystèmes et de la biodiversité, et soutient un développement rural inclusif

Sur 5,8 milliards d'euros de soutien financier que nous avons engagés pour des projets agricoles à destination des pays éligibles entre 2009 et 2018, seuls 13 % soutenaient exclusivement des projets agroécologiques, contre 24 % à destination de projets d'agriculture intensive, dont certains sont des mégaprojets agro-industriels. La prise en compte des objectifs climatiques est quasi absente. Sur les dix dernières années, seulement 1,4 % de nos financements au secteur agricole ont intégré ces objectifs climatiques. Pour illustrer ces chiffres, prenons le cas de la République démocratique du Congo (RDC), exemple frappant des incohérences de notre politique publique. Parallèlement à tous les projets de l'AFD destinés à soutenir les populations de la RDC,

Ce projet Feronia cumule toutes les dérives que permettent nos financements français à l'étranger : insuffisamment cohérents, insuffisamment contrôlés, insuffisamment « redevables ». En d'autres termes, ils défont d'une main ce qui a été fait de l'autre. fait de l'autre. Intégrer les politiques agricoles alimentaires dans la recherche de cohérence des politiques publiques ayant un impact sur les ODD n'est pas superflu. Pour le coup, c'est même une nécessité impérieuse.

Cet amendement vise à affecter au moins 50 % de l'APD aux services sociaux de base. En 2018, la France consacrait moins de 20 % de son APD totale aux services sociaux de base, tels que la santé, l'éducation, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, ou encore les systèmes de protection sociale. Déjà dans le monde pré-covid, nous n'étions pourtant pas sur la bonne voie pour atteindre les cibles fixées pour 2030 par l'Agenda des objectifs de développement durable. Puis, partout, la crise sanitaire et économique a révélé et exacerbé les inégalités d'accès à ces services, pourtant essentiels. La pandémie a mis en lumière le manque de financement chronique dont ils pâtissent, un désinvestissement qui dure depuis plusieurs décennies. Ces services sociaux de base constituent pourtant le socle de la réalisation des droits humains fondamentaux et la clé de voûte de la réduction de la pauvreté et des inégalités, notamment de genre. La pandémie a fait reculer radicalement l'accès à ces services, notamment dans les pays les plus pauvres et pour les populations les plus vulnérables et minorisées, au premier rang desquelles les femmes, les adolescentes et les filles. Pour la première fois depuis plus de vingt ans, l'extrême pauvreté va augmenter et les études démontrent que ce sont les plus pauvres qui s'appauvrissent encore. Ainsi, l'Afrique subsaharienne qui comptait déjà des taux de pauvreté élevés devrait abriter près d'un tiers des personnes nouvellement appauvries par la covid-19. Comme nous le soulignions précédemment, ce projet de loi doit traduire un engagement plus résolu et plus concret en la matière. C'est pourquoi nous proposons, par cet amendement, un fléchage d'une part importante de l'APD en direction des services sociaux

pour ce qui concerne la France ne nous permettra absolument pas d'atteindre les objectifs fixés par l'ONU. Il y a six ans, l'ONU adoptait l'objectif « Faim zéro » dans le cadre de l'Agenda 2030. L'objectif est de tendre à l'éradication de la sous-nutrition et de la malnutrition d'ici à 2030 en s'appuyant sur tous les leviers : lutte climatique pour enrayer le phénomène de stérilité des sols et l'impossibilité de faire pousser des productions, aide alimentaire, aide à la structuration des filières agricoles, mais aussi pacification du monde. Car, il faut le rappeler, les conflits sont directement responsables de plus de la moitié des crises alimentaires. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, au Yémen, près de 13,5 millions de personnes, soit environ 45 % de la population, sont dans une situation de crise alimentaire aiguë.

par la sous-nutrition d'ici à 2030. En intégrant dans les calculs les phénomènes de malnutrition, la FAO estime que 2 milliards de personnes sont dans une situation de précarité alimentaire. Ce constat, dramatique humainement, est d'autant plus insupportable que la production mondiale de nourriture est amplement suffisante pour nourrir tout le monde, et convenablement. La crise sanitaire n'a fait qu'exacerber une problématique déjà très lourdement présente. Le rapport d'Oxfam intitulé révèle que la famine a a concerné 121 millions de personnes supplémentaires en 2020, à la suite notamment de la disparition de l'équivalent de 305 millions d'emplois à plein temps selon

du Gouvernement ? La lutte contre les maladies et le soutien au système de santé constituent une priorité de la politique de développement de la France, comme le rappelle le rapport annexé au projet de loi.

consacre dès à présent 55 % de l'APD bilatérale en 2019, soit 4,7 milliards d'euros. Dans le cadre de l'APD « santé », la France a par ailleurs consacré

Mme Claudine Lepage. Cet amendement vise, d'une part, à prévoir un objectif de 85 % d'APD bilatérale programmable française ayant l'égalité femmes-hommes pour objectif principal ou significatif et, d'autre part, à affirmer les nouvelles ambitions de l'APD « genre ». Il est motivé par plusieurs constats. Depuis 2019, la France porte publiquement une diplomatie féministe dans les différents internationaux qui, pour l'instant, ne va pas de pair avec une véritable APD féministe. Le rapport de l'OCDE, de mars 2021 confirme la place de la France parmi les cinq derniers pays donateurs d'APD « genre

Égalité sur les droits des femmes, ce texte offre une occasion incontournable de s'assurer que la France passe des paroles aux actes et montre la voie d'une diplomatie féministe ambitieuse. Le choix de la cible spécifique de 85 % n'est pas anodin : d'une part, dans les intentions, il vise à harmoniser l'objectif français avec celui du plan d'action sur l'égalité des genres 2021-2025 de l'Union européenne ; d'autre part, dans la pratique,

Le même objectif à horizon 2025 est repris et recommandé par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes dans son évaluation de la diplomatie féministe française, avec un seuil intermédiaire de 60 % d'aide genrée d'ici à 2022.

Les projets sont ainsi marqués CAD 1 s'ils ont pour objectif significatif l'égalité et CAD 2 si l'égalité correspond à leur objectif principal. Le présent amendement vise à ce que la France se fixe un objectif pour 2025 de 20 % de projets soutenus ayant l'égalité femmes-hommes comme objectif principal.

française par l'objectif englobant de 30 % d'aide publique au développement de la France allouée aux 19 pays pauvres prioritaires. L'ensemble de ces pays ne reçoit que 15 % de l'aide française, un montant bien insuffisant pour retranscrire cette volonté de priorisation. De plus, sur les cinq premiers pays bénéficiaires de l'aide française, aucun n'appartient à la catégorie des pays les moins avancés ni ne fait partie des pays prioritaires. La qualité de l'APD dans la lutte contre l'extrême pauvreté va de pair avec un ciblage efficace vers les pays et les populations qui en ont le plus besoin. Or, sur le ciblage géographique, l'aide française souffre encore d'une forte dispersion et ne réserve pas de priorité aux pays les moins avancés, qui concentrent pourtant les poches d'extrême pauvreté dans le monde. L'alinéa 37 du rapport annexé au projet de loi prévoit que la zone Afrique et Méditerranée reçoive 75 % de l'effort financier de l'État et 85 % de celui de l'AFD, ce qui recouvre les subventions, mais aussi les prêts concessionnels. Sans grande différence avec la cible de 2014 qui plaçait l'effort financier de l'État à 85 %, est géographiquement trop large, car il inclut un grand nombre de pays à revenus intermédiaires au lieu de cibler les pays les moins avancés. Nous voulons donc remédier à cette situation et renforcer le ciblage de l'aide en direction des pays prioritaires.

Le cadre de partenariat global prévoit déjà que les 19 pays prioritaires bénéficient de la moitié de l'aide-projet mise en oeuvre par l'État, dont un tiers est concentré sur les pays du G5 Sahel. Par ailleurs, les deux tiers des subventions mises en oeuvre par l'AFD y sont consacrés. La cible proposée pourrait conduire à des effets pervers,

En 2018, selon l'OCDE, l'aide française se concentrait majoritairement sur des pays à revenus intermédiaires qui sont par ordre d'importance : la Colombie, l'Indonésie, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Cameroun, l'Inde, la Turquie, le Sénégal, l'Égypte et la Chine. Un seul pays parmi ces derniers appartient à la liste des 19 pays prioritaires. Il s'agit de remédier à cette situation afin d'assurer une plus grande efficacité de l'aide aux pays les plus pauvres, priorité de l'APD française.

Ce sujet, qui est au coeur de nos préoccupations à tous, doit figurer comme un élément essentiel de la réciprocité que nous attendons. S'il y a une seule référence à citer, c'est bien celle-là.

M. Thierry Cozic. L'alinéa 41 dresse une liste des questions sur lesquelles il est nécessaire d'accroître les synergies, en d'autres termes d'appliquer une approche transversale. Étonnamment, il manque un certain nombre de questions. La première est celle des inégalités sociales, qui relèvent d'une approche en matière d'éducation, de genre, d'accès aux infrastructures et d'insertion économique, pour ne citer que ces domaines. touche à l'urbanisation et relève tant du maintien du tissu économique et social en zone rurale, afin d'éviter l'exode rural et une urbanisation galopante qui accroît la pauvreté, que du développement durable, en promouvant des logements abordables et durables par exemple. La troisième a trait aux enjeux de diversité culturelle, qui concernent l'approche par le genre et la construction d'un développement au travers d'un dialogue entre les communautés et les ethnies. Cet amendement vise à remédier à ces manques.

explication de vote. Je saisis cette occasion pour revenir sur le volet urbanisation, notamment sur le logement social. J'ai déposé un amendement visant à instituer un dispositif de financement innovant supplémentaire reposant sur l'initiative des collectivités territoriales. Il s'agissait de créer un dispositif d'aide au logement abordable et durable dans le cadre de la solidarité internationale, en autorisant les collectivités territoriales, ainsi que les bailleurs sociaux français qui leur sont rattachés, sur la stricte base du volontariat des actions de coopération et de solidarité internationales conduites avec leurs homologues dans les pays éligibles compétents en matière de logement, dans le cadre d'un financement librement décidé par chaque collectivité. Cette mesure présentait un double avantage. D'une part, l'apport supplémentaire de financement contribuait à atteindre l'objectif de développement durable 11 qui vise, d'ici à 2030, à assurer l'accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs à un coût abordable, et à assainir les quartiers taudis. D'autre part, la création d'un nouvel axe de coopération dans le domaine du logement social aurait contribué à renforcer la qualité des politiques d'APD en la matière, à partir d'initiatives territoriales.

Mme Nicole Duranton. Lors de l'examen du texte en séance, les députés ont adopté un amendement visant à concrétiser la résolution n° 514 de l'Assemblée nationale pour la création d'une communauté méditerranéenne des énergies renouvelables. Les auteurs de cet amendement se félicitent d'un tel ajout et proposent de le compléter par une référence à l'action des collectivités territoriales, fortement impliquées dans la coopération portant sur le pourtour méditerranéen, et notamment la préparation du futur Forum de la Méditerranée.

au titre des priorités transversales l'engagement de la France à mettre en oeuvre le règlement européen relatif aux minerais dits « de conflit ». Il vise à conforter l'exigence de vigilance qui doit imprimer sa marque à ce projet de loi.

L'objet de ce règlement européen est d'empêcher l'importation de métaux et de minerais dits « de conflit » ayant contribué au financement de conflits armés ou à des atteintes aux droits de l'homme. Il est lié aux obligations européennes existantes en matière de devoir de vigilance à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importations d'étain, de tantale, de tungstène et d'or provenant de zones de conflit ou à haut risque. L'introduction de ces obligations à l'alinéa 45 du cadre de partenariat global apparaît ainsi justifiée.

Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement, qui non seulement singularise un règlement européen, mais

» de l'AFD, qui a été présenté à son conseil d'administration, détaille le bilan de l'Agence à l'égard de cet engagement que le ministère de l'Europe et des affaires étrangères considère comme rempli. Les auteurs de cet amendement saluent un tel engagement ambitieux et inédit en faveur du climat, qui honore la France. Avec cet amendement de précision rédactionnelle, ils soulignent que cet engagement doit être maintenu dans la durée et que le niveau d'exigence pourrait être rehaussé à l'avenir.

Il s'agit d'un amendement de reformulation et de précision de l'alinéa 47 existant. L'amendement vise d'abord à corriger la période de la septième reconstitution des ressources du Fonds pour l'environnement mondial (FEM),

le Fonds multilatéral pour la mise en oeuvre du protocole de Montréal (FMPM) à l'alinéa 47, qui liste tous les dispositifs multilatéraux pour le climat et l'environnement auxquels participe la France. Or chacun sait

fluides de remplacement de substances appauvrissant la couche d'ozone qui ont un fort potentiel de réchauffement climatique. Je souhaite que l'on puisse inscrire ce fonds multilatéral dans la liste, la France étant le quatrième contributeur à ce fonds sur la période de reconstitution 2018-2020.

à ce que, d'ici à 2030, 30 % de ses financements bilatéraux consacrés au climat présentent des cobénéfices pour la biodiversité. Dans ce contexte, nous proposons de renforcer les dispositions du cadre de partenariat global relatives à la biodiversité.

Il vise à corriger l'incohérence relevée entre les engagements de la France pour la biodiversité, pris lors des grands rendez-vous internationaux pour la planète, et la programmation des moyens financiers qui lui sont consacrés dans le cadre de ce

des moyens financiers consacrés à cette convergence. C'est pourquoi nous proposons logiquement de fixer à 800 millions d'euros le montant de cet accroissement pour augmenter les financements annuels favorables à la biodiversité de 1 milliard d'euros en 2019 avec un objectif de 1,8 milliard d'euros en 2025. Quel

Sur ce sujet, il convient d'interroger le Gouvernement sur l'état exact de nos engagements et sur la cohérence du montant affiché. Nous souhaitons

du changement climatique. Elle s'est engagée à faire de la biodiversité une priorité de son action diplomatique et l'a placée en haut de l'agenda international, en vue d'obtenir un résultat ambitieux lors de la COP 15 d'octobre 2021. À l'occasion du sommet de janvier 2021, des engagements déterminants ont été pris afin de promouvoir la convergence des financements climat et biodiversité. Il n'est toutefois pas possible d'inscrire dans la loi une nouvelle cible en volume sur l'APD en faveur de la lutte contre le changement climatique et de la protection de la biodiversité. Il serait tout aussi

Le présent amendement a pour objet d'assurer le respect du droit au consentement libre, informé et préalable des peuples autochtones dans les projets financés au titre de l'aide publique, en particulier concernant les projets de conservation de la nature et de la biodiversité. Aujourd'hui, 80 % de la biodiversité mondiale se situe dans les territoires des peuples autochtones. Les projets de protection de la biodiversité, comme les aires naturelles protégées, ne peuvent donc, en aucun cas, laisser de côté ces peuples dans la création et la gestion des projets d'aires protégées, protégées, qui mènent fréquemment à l'évacuation des habitants de ces territoires, malheureusement trop souvent en recourant à la violence. Pourtant, les agences et les organisations d'aide au développement ont tout intérêt à associer les peuples autochtones aux projets de protection de la diversité. C'est également ce qu'a démontré l'AFD dans un projet mené au Brésil, dans l'État du Mato Grosso, pour la protection de l'Amazonie. Un responsable d'équipe projet à la division agriculture et biodiversité de l'AFD a déclaré à ce sujet que soutenir les activités des peuples autochtones va contribuer justement à la sauvegarde de ces terres. Le constat fait par l'AFD est éclairant : « Les zones forestières situées en territoires indigènes sont celles où la déforestation progresse le moins ... pour peu que les populations aient suffisamment de moyens de contrôle. » Aussi, associer systématiquement les peuples autochtones au projet de l'AFD, lorsqu'ils sont concernés, passe nécessairement par l'assurance que leur consentement est pris en compte. Le contrôle systématique de cette prise en compte n'est pas une garantie superflue, car les populations autochtones, de par leur mode de vie en marge des institutions officielles et leur absence fréquente de représentation politique, n'ont, bien sûr, pas les moyens de défendre leurs intérêts auprès des autorités. Cet amendement vise donc à préciser que le respect du consentement de ces peuples vaut pour

monsieur le ministre,

M. Thierry Cozic. Cet amendement vise à compléter l'engagement de la France dans la lutte contre le trafic des espèces sauvages en promouvant la protection des espèces mentionnées dans la convention de Washington. En effet, le cadre de partenariat global fixe comme priorité transversale la nécessité de relever les défis environnementaux. Pour éviter la disparition de plus de 3 000 espèces animales et de plus de 40 000 espèces végétales, la France est signataire de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Quelque 182 pays sont signataires de cette convention et s'engagent à la respecter. Adopter cet amendement permettrait d'inscrire dans cette loi le texte de référence dans la lutte contre le braconnage et pour la sauvegarde de toutes les espèces. Enfin, cet amendement permet de garantir la biodiversité en renvoyant à un texte international de référence et renforce l'objectif premier de l'APD, fixé dans le cadre de la loi.

des adolescentes et des femmes fait partie intégrante du socle fondamental du développement durable, aux côtés de l'autonomisation politique, économique et sociale des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Selon le dernier rapport annuel du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), intitulé et publié le 14 avril 2021 dans 57 pays à travers le monde, près d'une femme sur deux voit son autonomie corporelle bafouée. Ces femmes se retrouvent ainsi privées de la possibilité de prendre leurs propres décisions sans crainte de subir des violences, qu'il s'agisse de relations sexuelles, du recours à la contraception ou encore de la recherche de soins de santé. de santé. Le constat de ce premier rapport des Nations unies est cinglant sur la capacité et les moyens des individus de faire des choix concernant leur corps. En somme, des centaines de millions de filles, d'adolescentes et de femmes sont victimes d'atteintes à leur autonomie corporelle, allant du viol à la stérilisation forcée, en passant par l'imposition de tests de virginité et de mutilations génitales. L'autonomie corporelle n'est pas seulement un droit, elle est le fondement même des autres droits humains. Elle est incluse, implicitement ou explicitement, dans de nombreux instruments internationaux relatifs aux droits humains.

de lever les obstacles à l'autonomisation et à l'émancipation des femmes. Pour que cette volonté politique se matérialise dans les faits, il est impératif de donner aux jeunes filles les clés nécessaires de cette émancipation dans les sphères sociale, économique et politique, notamment par la scolarisation et l'insertion professionnelle. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le présent amendement qui soutient la scolarisation des jeunes femmes. De nombreuses jeunes filles et femmes sont en dehors du système éducatif, et ce sont les mêmes que l'on retrouve massivement dans le secteur informel. L'informalité détériore les conditions de vie de ces femmes qui sont plus vulnérables et demeurent enfermées dans la pauvreté. Comme l'a rappelé Claudine Lepage, la pandémie de covid-19 a encore davantage fragilisé ces travailleuses. davantage fragilisé ces travailleuses. Si le genre est une variable déterminante, le niveau d'éducation l'est tout autant, puisque les risques d'occuper un emploi informel augmentent selon le niveau d'éducation. Or les jeunes filles et les femmes sont celles qui souffrent le plus d'un accès limité à l'éducation. Il est donc tout aussi important d'apporter un soutien aux structures associatives de terrain qui accompagnent au quotidien leur transition du secteur professionnel informel au secteur formel. Cela n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui ; en effet, en pratique, l'Agence française de développement soutient majoritairement des projets de grande envergure au détriment de ceux qui sont nés d'initiatives locales à la rentabilité moindre, puisqu'ils sont individuels. Pourtant, le contexte mondial nous démontre encore aujourd'hui l'importance de s'appuyer sur les acteurs associatifs. Je vous invite donc à voter cet amendement qui met l'accent

et soutient pleinement les efforts des Nations unies pour les déployer à tous les niveaux, en particulier dans les processus de paix. Si beaucoup de choses ont été réalisées depuis l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité, les auteurs de cet amendement estiment que beaucoup peut encore être fait. De même, ils jugent essentiel que la France continue à soutenir la mise en oeuvre de la résolution 2538 du Conseil de sécurité, adoptée à l'unanimité en août 2020, sur les femmes dans les opérations de maintien de la paix. Il convient de souligner qu'il s'agit de la première résolution autonome sur les femmes dans le maintien de la paix.

Le sport constitue un accélérateur de ces évolutions qu'il serait contre-productif de délaisser. C'est pourquoi cet amendement vient préciser le rôle du sport dans le soutien à l'égalité femmes-hommes.

Annoncée en 2019 par le Président de la République, la création du Fonds de soutien aux organisations féministes vise à soutenir les organisations féministes de la société civile opérant dans les pays partenaires de la politique de développement de la France. Copiloté par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères et l'AFD, ce fonds s'inscrit dans le cadre de la diplomatie féministe française et de la stratégie internationale de la France pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2018-2022. Il doit mobiliser 120 millions d'euros sur trois ans- 2020 à 2022 -et constitue un des « livrables » de la France pour le forum « Génération égalité » qui doit se tenir au mois de juillet prochain.

Ses modalités sont également innovantes du fait de la souplesse de son fonctionnement et la complémentarité de ses trois canaux de financement. Innovation et traduction pure et simple des engagements français en matière de diplomatie féministe et de rapprochement avec la société civile, ce fonds doit être valorisé dans le temps long et pérennisé.

de la politique diplomatique féministe de la France. Au vu de la priorité annoncée dès l'article 1 A en matière de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et les filles et les garçons, il semble incohérent de ne pas mentionner le Fonds de soutien aux organisations féministes dans le cadre de partenariat global. Par ailleurs, monsieur le ministre, une pérennisation de ce fonds au-delà de 2022 est-elle envisagée ? Cela semble, aujourd'hui, plus encore nécessaire qu'hier. Selon le dernier rapport du forum économique mondial de Davos, il faudra encore compter 135,6 années avant de parvenir à la parité à l'échelle mondiale, tant sur le plan économique que dans l'accès à la santé ou encore à l'éducation. Dans le domaine politique et la représentation législative et exécutive, la crise nous a fait reculer de cinquante ans, pour atteindre une parité Dans ce cadre, la mobilisation active des associations féministes dans les pays éligibles à l'APD est un levier précieux pour faire avancer la condition des femmes dans ces pays. La crise sanitaire et économique a encore fait reculer la cause des femmes à travers le monde, notamment en touchant plus fortement ces dernières. Selon les chiffres de l'Organisation internationale du travail, la perte d'emploi des femmes a atteint 5 % en 2020 contre 3,9 % chez les hommes, étude à l'appui. En parallèle, nous avons assisté à une aggravation de la double charge des femmes entre le travail et les responsabilités de la maison, avec les tâches ménagères, la garde des enfants et les soins aux personnes âgées qui leur incombent de manière disproportionnée. De plus, le dernier rapport d'ONU Femmes pointe une augmentation inquiétante des violences à l'égard des femmes, tout particulièrement la violence domestique intrafamiliale. Une nouvelle fois, ce sont bien souvent les organisations féministes de la société civile qui sont en première ligne pour prévenir et secourir les femmes victimes de violences. On assiste ainsi à un véritable recul des progrès faits en matière de droits des femmes ; il est donc nécessaire de soutenir plus massivement et de manière pérenne ces associations.

La diplomatie féministe ne peut s'affranchir de la participation des associations, des collectifs et des entités locales qui tentent de résorber les inégalités entre les hommes et les femmes dans leur propre pays. Nous devons donc soutenir ceux et celles qui, sur le terrain, oeuvrent à la défense de l'égalité dans des conditions souvent difficiles, particulièrement à l'heure à l'heure de la pandémie qui a creusé l'écart de pauvreté entre les hommes et les femmes. On estime ainsi que 47 millions de femmes et de filles supplémentaires vont basculer sous le seuil de l'extrême pauvreté entre 2019 et 2021, à l'heure où l'accès à l'éducation, à la contraception, à la santé et à un soutien psychologique et politique est souvent le fait d'associations locales qui se battent pour l'émancipation des femmes. C'est donc dans ce contexte que tous les pays se revendiquant d'une diplomatie féministe ont mis en place des fonds de soutien destinés aux organisations féministes. Le Canada, par exemple, s'est engagé à investir 300 millions de dollars dans son « Fonds égalité » à destination des organisations locales. La Suède investit 100 millions d'euros entre 2018 et 2022 dans son plan d'action pour une politique étrangère féministe, dont une large part est destinée au soutien des organisations locales féministes.

au-delà de 2022, en cohérence avec les nouvelles orientations du texte, qui s'étendent désormais à 2025, en cohérence avec les objectifs de la diplomatie féministe française. L'amendement

2 intitulée « Soutenir la grande cause du quinquennat qu'est l'égalité entre les femmes et les hommes et entre les filles et les garçons ». En effet, les filles demeurent un public vulnérable parmi les filles demeurent un public vulnérable parmi les vulnérables et se trouvent encore trop souvent négligées sur les plans de la santé, de l'éducation, de la nutrition et de la protection. Une mobilisation forte et marquée est donc indispensable. L'égalité filles-garçons est une condition incontournable à la réalisation de l'égalité femmes-hommes dont le Gouvernement a fait une grande cause du quinquennat. L'égalité filles-garçons s'inscrit dans un continuum avec l'égalité femmes-hommes qu'il est important de rappeler dans ce texte pour qu'il soit considéré dans l'ensemble des programmes, de façon intégrée et transversale.

Mme Claudine Lepage. Le cadre de partenariat global permet de fixer des objectifs à l'horizon de 2025. Dans le cadre du marquage « égalité femmes-hommes », il est important que la France se fixe des objectifs ambitieux si notre pays veut être à la hauteur des enjeux. La diplomatie féministe doit avoir des instruments pour assurer son application. Le marquage « genre » des projets soutenus par le biais de notre aide publique au développement en est

Cet amendement vise à les nommer expressément dans le cadre de partenariat global. Il convient de ne pas se limiter aux « déterminants de la fécondité », expression qui ne prend en compte que la dimension reproductive de la sexualité. En vertu de ce que l'on appelle « les droits sexuels et reproductifs », chacun devrait avoir le droit de choisir son partenaire, son mode de vie, de se marier ou non, d'avoir ou non des enfants ... Ces choix doivent pouvoir être assumés librement, sans contrainte

des genres 2021-2025 de l'Union européenne, dont la feuille de route a été dévoilée en mars 2020, aligne l'action de l'Union européenne sur les engagements internationaux, en particulier dans le cadre de la stratégie de Lisbonne de 2000. Ainsi, il s'appuie sur l'Agenda 2030 des Nations unies sur le développement durable, la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, d'action de Pékin des Nations unies d'action pour la promotion des droits des femmes et le programme des Nations unies pour les femmes, la paix et la sécurité. Ce plan reconnaît que, pour faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, il faudra des politiques de transformation, des changements systémiques et un engagement politique.

Une telle réaffirmation nous paraît nécessaire compte tenu des observations de la Cour des comptes sur la stratégie 3D- défense, diplomatie, développement -de la France au Sahel. la Cour des comptes souligne que, si les dépenses françaises ont plus que doublé entre 2012 et 2018, passant de 580 millions à 1,35 milliard d'euros, la majorité de ces sommes concernent des dépenses militaires. L'aide publique au développement n'a pas suivi la même progression. Les complémentarités entre les actions militaires et civiles d'aide à la stabilisation et au développement doivent être recherchées et se traduire dans l'organisation de la réponse française, notamment avec une coopération interministérielle renforcée. L'alinéa 57 doit aussi réaffirmer des principes guidant l'action humanitaire et la gestion de crises, en cohérence avec notre défense du principe de non-discrimination de l'aide. Ce n'est pas inutile au regard de la multiplication des « zones grises » où se mêlent populations et combattants.

l'alinéa 58, qui prévoit que la France promeut une approche globale des fragilités et des crises pour mieux coordonner tous les acteurs du développement et de l'humanitaire, et, surtout, par l'alinéa 59,

de la France représente un pilier de notre politique étrangère et de développement, comme je l'ai indiqué dans mon propos introductif. Je veux d'ailleurs, à cet égard, redire devant votre assemblée l'importance de notre engagement humanitaire.

dont l'objectif est de « promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous ». Il paraît important de faire « paix », laquelle est structurante dans l'Agenda 2030, qui s'organise autour de la planète, des populations, de la prospérité, de la paix et des partenariats.

dont la France est partie prenante et dont l'un des objectifs est de « promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous

L'aide publique au développement ne devrait pas être détournée pour des objectifs étrangers au développement. Elle devrait être entièrement dévolue au soutien des populations. Notre devoir envers celles-ci est de faire en sorte qu'elles vivent en paix et non pas seulement en sécurité, notion qui, au-delà d'une possible ambiguïté, ne couvre tout simplement pas les exigences de la paix. Nous proposons d'être plus ambitieux envers les populations que nous soutenons et d'orienter les politiques publiques vers un effort de paix, de justice et de construction d'institutions protectrices. La parole est à Mme Claudine Lepage, pour

On le sait, le développement contribue à la création d'un environnement propice à la sécurité et au renforcement de l'État de droit et, inversement, les gains en matière de sécurité assoient les conditions d'un développement durable en en faveur des populations. Grâce à la reconnaissance de ce lien entre sécurité et développement, la France peut engager le processus de réforme des systèmes de sécurité, dont le but est de renforcer

en général. À titre d'exemple, sur les 258 millions d'enfants et d'adolescents qui n'avaient pas accès à l'école en 2018, près de 130 millions sont des filles âgées de 6 ans à 17 ans, dont 75 % d'adolescentes. Par ailleurs, au moins 200 millions de filles et de femmes en vie aujourd'hui ont subi des mutilations génitales dans trente pays, et 12 millions de filles sont mariées de force chaque année.

... Partout dans le monde, les filles demeurent un public particulièrement vulnérable, dont la situation spécifique doit absolument être prise en compte dans le cadre d'une diplomatie féministe cohérente.

Ainsi, près de 12 millions de filles sont mariées de force chaque année, et même une fille sur trois dans certains pays. On prédit que 10 millions de filles supplémentaires seront exposées au mariage forcé en conséquence de la crise du covid-19 et du fait de la déscolarisation.

dans certains pays. La situation actuelle est particulièrement dramatique, car l'on estime que la pandémie pourrait entraîner, au cours des dix prochaines années, 2 millions de cas de mutilations génitales féminines qui auraient été évitées en temps normal. La protection des filles est donc un enjeu fondamental de la diplomatie féministe, que nous devons réaffirmer dans ce contexte préoccupant. Leur situation particulière doit être mentionnée dans le projet de loi. À cet égard, constitue une précision indispensable pour orienter une mobilisation forte des politiques publiques de développement à leur profit. La parole

Elle agit comme un facteur de protection : le maintien à l'école ou même la préservation d'une éducation informelle permettent, par exemple, d'éviter le travail des enfants ou le mariage des filles. L'éducation est donc un droit et un besoin fondamental, autant qu'un levier pour préserver les enfants dans les crises.

grâce à un cadrage législatif clair et précis. L'école est un moteur de droit. Nous ne pouvons pas oublier l'importance de l'éducation pour l'émancipation collective et individuelle, la construction et la reconstruction de soi et, enfin, le développement dans tous les pays du monde.